Sur la forme, les parlementaires de la majorité sénatoriale n'ont eu de cesse, comme le Gouvernement d'ailleurs, de répéter que l'examen de ce projet de loi ne devait pas être l'occasion de débattre de la GPA.

Pourquoi une telle incohérence et un tel acharnement à priver des enfants de filiation ? C'est de l'intérêt supérieur d'enfants français nés hors de France qu'il s'agit, de leur droit à avoir une filiation établie en conformité avec nos exigences conventionnelles et selon la force probante que donne actuellement l'article 47 de notre code civil aux actes de naissance étrangers.

Comment cautionner ces atteintes portées aux droits de l'enfant au seul motif d'un désaccord avec des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, au contraire, devraient être saluées au nom de l'intérêt de l'enfant ?

Cet article 4 est inadmissible et indigne de notre assemblée, en ce qu'il s'inscrit en contradiction profonde avec l'intérêt de l'enfant.

la filiation qui peut être établie est en général la filiation paternelle, quand le père est l'auteur des gamètes ayant permis

Par conséquent, on ne prive pas l'enfant d'une filiation à laquelle il aurait droit en refusant de transcrire dans les actes d'état civil français une filiation maternelle

c'est rappeler que la transcription à l'état civil français est bien sûr possible, mais dans la limite où elle correspond à la vérité de la filiation,

Le président Retailleau et plusieurs de ses collègues en ont décidé autrement, et nous allons donc en débattre. Nous parlons de quelques centaines d'enfants, nés dans le cadre d'un processus aujourd'hui illégal en France

nouvelle, puisque l'assemblée plénière de la Cour de cassation puis la première chambre ont toutes deux, voilà seulement quelques semaines, pris la décision

collègues : « Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France, mais je m'engage à ce que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue par l'état civil français. Comme tous les enfants, nous avons le devoir de les protéger. La circulaire du 25 janvier 2013 permettant de reconnaître les enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger n'est pas uniformément appliquée sur le territoire français, ni dans tous les consulats. Je souhaite donc la compléter selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Si, en droit français, les conventions de GPA sont interdites, cet amendement vise néanmoins à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'est pas responsable de son mode de procréation. de garantir le respect du principe d'égalité des enfants devant la loi, en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, s'appuyant sur l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 avril 2019. En effet, notre haute juridiction vient d'étendre sa jurisprudence du 4 octobre 2019 en ordonnant, par une série de quatre arrêts rendus en décembre dernier, la transcription totale dans l'état civil français de l'acte de naissance étranger, indépendamment du mode de conception de l'enfant. La Cour de cassation a donc contredit la cour d'appel de Rennes, qui avait admis la transcription partielle d'actes de naissance étrangers en ce qu'ils désignaient le père biologique d'une GPA, mais avait refusé cette transcription en ce qu'ils désignaient le « père d'intention La Cour de cassation prend donc ses distances avec une conception purement biologique de la filiation. Les parents de même sexe d'un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée peuvent demander la transcription totale de l'acte d'état civil étranger, s'il est conforme au droit local. Ainsi, en cas de GPA pratiquée légalement à l'étranger, le père d'intention n'a plus à engager une procédure d'adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse. Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d'obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu'elle a été établie dans l'État de naissance de ces enfants. Le dispositif maintient toutefois le contrôle que l'État français est en droit d'exercer sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l'absence de violation, par ce jugement, de l'ordre public international français et de l'absence de fraude.

Par une circulaire de la garde des sceaux en date du 29 janvier 2013, il est permis d'inscrire aux registres d'état civil français les enfants nés à l'étranger Cette circulaire a, depuis, été validée par le Conseil d'État, en 2014, et a ouvert la voie à une jurisprudence solide du tribunal de grande instance de Paris. J'ai bien évidemment toujours été favorable à ces décisions de justice, estimant que les enfants nés de GPA n'avaient pas à être punis pour les actes illégaux de leurs parents.

par ces décisions de justice, afin de garantir une véritable sécurité juridique pour les nouveau-nés fruits d'un contrat de gestation pour le compte d'autrui conclu à l'étranger. J'entends évidemment les réticences de nos collègues de tous bords politiques tenant au risque de marchandisation du corps des femmes en situation de précarité si cette pratique n'était pas éthiquement encadrée.

peut nous rassembler toutes et tous. bien même cette pratique reste interdite en France depuis la loi du 29 juillet 1994. C'est un état de fait que nous devons prendre en compte dans notre travail législatif. Environ 2 000 enfants seraient concernés.

si le code civil dispose explicitement que toute convention ayant pour objet une gestation pour autrui est nulle, le législateur de 1994 n'a pas prévu de solution de droit pour les enfants nés à l'étranger en violation de cette interdiction. Or ces

L'amendement de notre collègue Bruno Retailleau introduit une disposition visant à clarifier cette situation, en prévoyant que, pour le parent d'intention, l'adoption doit rester la seule voie administrative et judiciaire possible pour établir un lien de filiation avec l'enfant. C'est justement ce qu'ont contesté les époux

a une incidence sur l'établissement de la nationalité des enfants. Nous proposons donc de modifier le dispositif de l'article, afin de permettre la transcription des actes d'état civil étrangers un juge, solution plus satisfaisante du point de vue de l'intérêt supérieur des enfants concernés.

comme cela se fait actuellement dans les consulats, en cas de naissance d'enfants français à l'étranger. Les auteurs de l'amendement n'entendent pas remettre en cause l'interdiction de la GPA en France, mais ils considèrent que, en matière de procréation et de filiation, il est illusoire de considérer que l'établissement de longs parcours administratifs et judiciaires permettra de lutter contre le recours à cette pratique à l'étranger. Dans l'intérêt des enfants concernés, il est donc proposé de simplifier ces procédures, tout en prévoyant quelques garanties protectrices pour les mères porteuses et les mineurs. En conclusion, je voudrais remercier M. le président de la

La France a fait le choix d'interdire la GPA, au nom de principes éthiques sur lesquels il n'est pas question de céder. Il existe cependant une réalité : nos frontières sont ouvertes et des couples se rendent à l'étranger pour obtenir un enfant par le biais d'une GPA. Nier cette réalité pourrait conduire à pénaliser des enfants en raison de choix effectués par leurs parents. Il convient donc de trouver un équilibre entre l'effectivité de l'interdiction de la GPA et le droit, pour les enfants, à avoir un état civil et une vie familiale normale. Il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que, lorsqu'un couple avait eu recours à une GPA à l'étranger,

Le Gouvernement approuvait et approuve toujours cet équilibre, qui permet à la fois un contrôle du juge français sur les GPA réalisées à l'étranger et une protection des intérêts et des droits en présence, notamment, bien sûr, ceux de l'enfant.

l'homme par un avis du 10 avril 2019 précisant que la jurisprudence de la Cour de cassation était compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH a posé des conditions relatives à l'accès à la procédure d'adoption, mais, en décembre dernier, elle a redit que la procédure d'adoption française permettait de donner aux enfants nés d'une GPA à l'étranger une filiation dans des conditions conformes à la jurisprudence et aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le 18 décembre dernier, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure, en permettant la transcription de plein droit des actes de naissance établis à l'étranger sans passer par l'adoption. Techniquement, la Cour de cassation a modifié son interprétation de l'article 47 du code civil sur la régularité des actes de l'état civil étranger.

Jusque-là, la Cour de cassation considérait que la « conformité à la réalité » s'appréciait au regard de la loi française. Pour la GPA, cela signifie que l'acte de naissance qui désigne la mère d'intention comme mère n'était pas conforme à la réalité, puisque, en droit français,

au regard non plus des critères de la loi française, mais des critères de la loi nationale étrangère. Évidemment, cela change les choses. Le Gouvernement ne peut se résoudre à ce nouvel état du droit, je le dis clairement. En il supprime notamment tout contrôle juridictionnel sur les GPA réalisées à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de revenir à la situation antérieure à cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Le passage par la procédure d'adoption me paraît indispensable en ce cas, car seule l'intervention du juge dans le cadre de la procédure d'adoption permet d'opérer un contrôle dans l'intérêt de l'enfant, notamment de s'assurer de l'absence de trafic d'enfants.

à l'article 47 du code civil, que la conformité de l'acte étranger s'apprécie au regard des critères de la loi française.

est soumise permet en effet de s'opposer à des transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d'autres raisons- on peut penser par exemple aux actes de naissance qui incluent plus de deux parents,

réalisée préalablement aux états généraux de la bioéthique et à la révision de la loi relative à la bioéthique, a indiqué clairement que la GPA heurte la substance même du modèle bioéthique français.

encore une fois, le principe de l'interdiction de la GPA en France. En outre, selon les dispositions de ces amendements, le procureur de la République serait tenu de procéder à la transcription du jugement sans aucun contrôle de fond sur le respect de l'intérêt de l'enfant, ce qui ne sera pas le cas si la procédure d'adoption est mise en oeuvre

qui reprend elle-même celle de la Cour européenne des droits de l'homme sur la filiation d'un enfant issu d'une gestation pour autrui. Cependant, les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont été établis non pas pour la France, mais pour l'ensemble des États, de sorte qu'ils sont relativement vagues

sauf s'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Vous souhaitez donc préciser que cette réalité doit être appréciée au regard de la loi française.

estimant que « le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l'état civil français pour autant qu'ils désignent la mère d'intention comme étant leur mère n'est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis ». Cela signifie

situation actuelle a conduit un certain nombre de parents à se tourner vers la CEDH et la Cour de cassation pour qu'elles établissent le droit de leur enfant à avoir un état civil français.

une femme seule ou un couple non marié. Mais la Cour de cassation, par son arrêt du 4 octobre 2019 et ses trois arrêts du 18 décembre 2019, a tranché dans l'intérêt de l'enfant.

qui devrait prévaloir dans notre système juridique -, en permettant désormais la transcription intégrale des actes de naissance des enfants français nés d'une GPA à l'étranger, mais la parole donnée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale semble remise en cause. Dans un souci de sécurité juridique, il convient donc d'apporter dans la loi les précisions nécessaires pour que tous les enfants aient les mêmes droits

Le mérite de la commission spéciale est d'avoir clairement donné un coup d'arrêt à cette exigence qui semblait grandir d'une transcription intégrale des actes d'état civil rédigés rédigés à l'étranger à la suite d'une gestation pour autrui. Qu'on reconnaisse que le père génétique est le père, c'est une chose qu'on donne au père d'intention ou à la mère d'intention un statut ou de père ou de mère, c'en est une autre. Il me semble que les amendements visant en réalité à consolider la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire tous,

que la réalité de la situation reconnue par l'acte d'état civil étranger doit être appréciée

et je ne vois pas comment la Cour de cassation pourrait s'appuyer sur cette mention pour renoncer à la nouvelle jurisprudence qu'elle vient d'esquisser. La commission spéciale, elle, a dit les choses nettement nettement : on doit continuer à transcrire partiellement les actes d'état civil, pour la filiation paternelle établie, et pas pour la filiation des parents d'intention.

française en difficulté par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme dans tous les cas où l'adoption par le parent d'intention n'est pas possible. La CEDH a jugé

a estimé que lorsque la filiation n'est plus possible, la transcription de l'acte de naissance étranger à l'égard du parent d'intention est la seule manière de reconnaître

à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n'est pas, monsieur le président Bas, purement cosmétique

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

les résultats du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

l'origine de l'introduction de cet article, de faire obstacle à une inflexion jurisprudentielle de la Cour de cassation qui, dans le cadre de son dialogue avec la Cour européenne des droits de l'homme et en réponse à différents cas, avait admis une transcription totale de l'acte de naissance lorsqu'elle était la solution possible dans l'intérêt de l'enfant ou lorsque l'acte de naissance établi à l'étranger était probant. Environ 2 000 enfants seraient concernés par une filiation partielle du fait de cette interdiction. Cette filiation partielle rendrait la situation de ces enfants plus vulnérable en cas de décès ou de défaillance du seul parent reconnu. Les auteurs du présent amendement estiment que, dans l'intérêt supérieur de l'enfant,

intention n'est pas de reconnaître un quelconque droit à la GPA ; notre droit interne est formel à ce sujet. Il s'agit de donner une identité pleine et entière à l'enfant. Gardons à l'esprit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer avant toute autre considération. La première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que la cour d'appel de Rennes en sont venues à la même conclusion : la transcription intégrale des actes de naissance est compatible avec le droit à la vie privée des enfants. Il serait en effet impensable de priver l'enfant de son état civil français et de sa stabilité administrative. Peu importent les choix des parents, l'enfant n'a pas à en subir les conséquences. L'administration française doit lui procurer un statut fixe, stable et juste. Il y va de ses légitimes droits fondamentaux. Interdire totalement l'établissement du lien de filiation entre un parent et son enfant biologique né d'une GPA à l'étranger est contraire au droit des enfants et au respect de leur vie privée, au sens de l'article 8 de la À deux reprises, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d'un enfant né par GPA à l'étranger. Les récentes décisions judiciaires vont dans le même sens. Il est temps de suivre la logique de nos juridictions et d'aligner la loi avec la jurisprudence en cours.

En tant que sénateur représentant les Français établis à l'étranger, je sais les difficultés déjà souvent rencontrées par nos compatriotes, selon leur pays de résidence, pour faire transcrire l'acte de naissance étranger de leur enfant. Je n'ose imaginer l'étendue des dégâts si cet amendement gouvernemental était adopté à l'Assemblée nationale Il est contraire à nos engagements conventionnels et à notre droit prétorien, en particulier à l'analyse faite de l'article 47 du code civil par le Conseil d'État dans l'arrêt du 31 juillet 2019. La réalité des faits déclarés dans l'acte étranger doit s'apprécier selon le droit local, et non selon le droit français. C'est ce qu'a décidé et précisé le Conseil d'État. C'est aussi ce que prévoient nos engagements conventionnels en matière d'actes d'état civil. Un tel bouleversement des règles relatives à l'état civil aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État et ne pas être introduit perfidement, par voie

De plus, comment exiger des autres États qu'ils reconnaissent les actes de naissance dressés en France pour leurs ressortissants nés dans notre pays si nous remettons systématiquement en cause les leurs au regard de la loi française ? Le Gouvernement n'a pas soumis son amendement au Conseil d'État. J'espère qu'il le fera avant la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale.

en accord avec le principe selon lequel le législateur doit reprendre la main sur cette question.

parent d'intention. Enfin, comme l'a jugé l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 octobre 2019, lorsque l'adoption n'est plus possible, la transcription de l'acte de naissance

à la traduction d'une recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur la création d'un statut du donneur d'organes. Il prévoit donc la création de ce statut, avec deux dimensions. Il s'agit d'abord de reconnaître et de valoriser donneur. Tous les acteurs que nous avons auditionnés, depuis l'Agence de la biomédecine jusqu'aux associations de patients et aux professionnels, nous ont indiqué que c'est un élément important pour favoriser le développement de la greffe dans notre pays.

: La parole est à M. Daniel Chasseing. Cet amendement a pour objet de garantir le droit à l'information des personnes en attente de greffe sur la qualité des greffons qui pourront leur être proposés, ainsi que sur leur droit de refus de certaines catégories de greffons, le cas échéant. Il vise aussi à confier à l'Agence de la biomédecine une mission d'information des publics, en particulier des patients concernés par la greffe. En effet, avec les progrès de la greffe, des organes qui autrefois pouvaient être exclus du prélèvement sont désormais transplantés. On parle de reins « à critères élargis » venant de donneurs donneurs « suboptimaux », par exemple des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies. On estime qu'environ la moitié des reins greffés sont désormais « à critères élargis ». Dans les faits, les patients sont très peu et mal informés sur la qualité du greffon qu'ils reçoivent.

leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus

est à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à prévenir d'éventuels dévoiements de la pratique du don d'organe, du côté tant des donneurs que des receveurs. En effet, l'article 5 prévoit d'étendre le don croisé d'organes à quatre paires de donneurs et receveurs tout en autorisant le recours, dans une chaîne de dons croisés, à un organe prélevé sur une personne décédée. Nous sommes bien évidemment favorables à une telle mesure, qui permettra de sauver des vies. Néanmoins, nous pensons que de telles procédures doivent être encadrées, tant l'enjeu est d'importance. le développement des réseaux de communication nous fait craindre l'établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l'encadrement établi pour le don d'organe entre personnes vivantes. Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d'anonymat et de gratuité du don. L'Agence de la biomédecine a établi, dans son bilan de 2017, que 23 828 personnes ont eu besoin d'une greffe, soit environ mille de plus qu'en 2016.

pourquoi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à près de 10 000 le nombre de transplantations illicites de rein réalisées chaque année, de 5 % à 10 % des transplantations effectuées dans le monde étant illégales. Le présent amendement a pour objet de garantir à tous les receveurs et potentiels receveurs, ainsi qu'aux donneurs, l'égalité de traitement qui leur est due, sans que des conditions économiques ou des privilèges induits par l'appartenance à des groupes de sociabilité dédiés

Le donneur est informé par un comité d'experts et doit exprimer son consentement au don devant un magistrat, afin d'éviter que sa décision résulte de pressions. Passer outre cette procédure est déjà réprimé par le code pénal. Les sanctions prévues sont lourdes : elles sont de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende pour « le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui ». Par ailleurs, la loi de bioéthique de 2011 a déjà confié à l'Agence de la biomédecine la mission de dresser, dans son rapport annuel,

le tourisme de transplantation, en informant les patients en attente d'une greffe des risques juridiques et médicaux que présente le recours à une greffe d'organe à l'étranger. Compte tenu de l'augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d'attente grandissantes, les Français qui ont besoin d'une greffe trouvent, grâce à la mondialisation et à internet, des solutions rapides et moins onéreuses. Ils peuvent aujourd'hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par internet. Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlé incontrôlé où le prélèvement d'organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques et où les citoyens français sont exposés à des risques sanitaires inconnus. Pour garantir un accès aux soins qui préserve la sécurité des malades et respecte les principes éthiques, il est essentiel que nos concitoyens soient sensibilisés aux risques sanitaires qu'ils encourraient

La formulation de votre amendement me semble un peu vague. Vous exprimez une intention, celle d'éviter le « tourisme de transplantation

Même avis ! la durée médiane d'attente, pour une greffe de rein, varie fortement selon l'établissement où les patients sont inscrits : un peu plus d'un an à Caen et plus de cinq ans à Paris ans à Paris en 2017. Il est proposé d'élever la lutte contre ces inégalités au rang de priorité nationale et de garantir que la répartition équitable des greffons à l'échelle nationale, de formaliser le processus d'élaboration et de modification permanente des règles de répartition, qui manque actuellement de transparence, et de transposer ces modifications dans les missions de l'Agence de la biomédecine, qui serait ainsi chargée de veiller au respect des bonnes pratiques. Quel est l'avis de

La loi affirme déjà depuis 2004 un principe d'équité dans les règles de répartition et d'attribution des greffons. Les échanges à ce sujet ont été nombreux. Je voudrais souligner que la composition du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui comprend notamment des représentants d'associations, permet de répondre à votre souhait que ces règles de répartition soient élaborées dans un cadre collectif et transparent. Je dois dire que je partage votre constat sur les marges de progrès dans la mise en oeuvre de ces principes par l'Agence de la biomédecine.

en effet essentiel de se prémunir contre le développement d'un marché de la transplantation, de protéger nos concitoyens des risques sanitaires qu'ils encourent en recourant à une transplantation à l'étranger. La mise en place d'un registre national de patients transplantés à l'étranger constituerait le moyen le plus efficace pour connaître la situation réelle du trafic d'organes impliquant des ressortissants français. Ce registre permettrait de recenser les informations relatives aux greffes d'organes réalisées à l'étranger, de mieux appréhender le phénomène du tourisme de transplantation, qui existe bel et bien, et d'améliorer la connaissance des profils des couples

ce cadre, l'Agence de la biomédecine procède à une enquête tous les deux ans, sur la base d'un questionnaire adressé aux équipes médicales de dialyse et de greffe rénale afin de recueillir des informations sur d'éventuels cas de greffes pratiquées à l'étranger.

être en mesure de connaître les personnes se faisant greffer à l'étranger. L'Agence de la biomédecine a la mission de rendre compte ; elle le fait avec célérité. Nous savons exactement,

présent amendement vise à garantir le droit à l'information, en prévoyant de formaliser dans le code de la santé publique l'obligation, pour les professionnels de santé chargés de patients dont l'évolution la maladie rénale pourrait nécessiter, dans un délai de deux ans, le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de greffe et de dialyse, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences.

Même avis.

dresse un bilan mitigé de la situation : « Le nombre de malades en attente d'un organe est près de quatre fois supérieur aux greffes réalisées et, dans le même temps, en moyenne 550 d'entre eux décèdent chaque année, depuis plusieurs années. Cet amendement vise à remédier à cet état de fait. Nous proposons d'ouvrir la possibilité, pour chaque assuré social, de faire figurer sur sa carte Vitale son accord au prélèvement d'organes à des fins de greffe en cas de décès.

Le rapport précise que les « dispositions trop peu connues, y compris des établissements de santé, induisent des démarches souvent complexes pour les donneurs ailleurs, l'une des conclusions de la mission sur le prélèvement d'organes du député Jean-Louis Touraine présentées le 20 décembre 2017 soulignait que le taux de refus important peut s'expliquer notamment par des « contextes défavorables qui mettent un coup d'arrêt à un prélèvement possible, le choc émotionnel subi par les familles l'emportant souvent sur la volonté du défunt. La médiation prévue dans notre amendement permettrait de respecter le choix de l'assuré tout en évitant de douloureux questionnements aux proches endeuillés. De plus, dans le cas où cette mesure serait adoptée, sa publicité permettrait une communication d'ampleur en direction du grand public, encore trop peu informé

En ce qui concerne la façon dont s'exprime le consentement au don d'organes, la loi de 2011 a prévu que les professionnels de santé

façon régulière. Toutefois, inscrire sur la carte Vitale l'expression du consentement de la personne reviendrait à renverser à nouveau le mode de consentement et induirait une confusion. Nous sommes dans la construction d'un mode de consentement ; celui-ci est imparfait, il doit progresser, nous en avons tous conscience, les professionnels et les associations de patients au premier chef, mais renverser le mode d'expression du consentement par l'inscription sur la carte Vitale d'un accord, donc revenir à une situation antérieure, serait

sauf inscription du refus sur le registre des refus de l'Agence de la biomédecine. Il est important de le souligner afin que nos concitoyens puissent se poser cette question en leur

à ce qu'est maintenant notre société ! Mes chers collègues, le modèle de la famille constituée d'un père et d'une mère a longtemps été la norme et est certes toujours fortement majoritaire, mais les familles se diversifient et le droit ne saurait exclure certaines d'entre elles. Les familles monoparentales et homoparentales existent également ; elles ne sont pas moins légales ni moins légitimes et leur existence mérite d'être validée dans nos textes juridiques. En effet, quand ces familles ne sont admises que dans les jurisprudences et restent ignorées par la plupart de nos textes de loi, nous perpétuons un environnement législatif discriminatoire à leur égard. Il est temps que le législateur se saisisse de cette question. Ainsi, dans un souci d'équité et d'uniformité, le présent amendement tend à remplacer toutes les occurrences, dans le code de la santé publique, des termes « père et mère » par le mot plus neutre de « parents ». Cette modification permettrait d'englober tous les types de familles qui existent dans notre société, afin de leur donner non seulement une existence juridique tangible, mais également une légitimité sociale. Quel est l'avis de

Ainsi, en matière d'aide sociale accordée aux étudiants et élèves sous forme de bourse d'études, il est accordé une majoration de points si « le père ou la mère » élève seul son enfant. La formulation n'a plus de sens si l'on remplace cette mention par « les parents